Composé à 92 % de PME qui investissent et innovent dans ce domaine hautement stratégique et compétitif, le secteur des dispositifs médicaux, marqué par une très forte hétérogénéité, est durement affecté par la crise sanitaire, en raison de la diminution nette des actes médicaux liée aux restrictions destinées à contrer la pandémie. Si la baisse de prix de 150 millions d'euros sur les dispositifs médicaux prévue dans le projet de loi obéit à une perspective légitime et nécessaire de rééquilibrage des dépenses publiques, elle ne saurait ignorer des considérations de politique industrielle devenues fondamentales pour notre souveraineté, notre compétitivité et l'emploi en France et dans l'Union européenne, dans un secteur hautement stratégique pour notre pays et bouleversé par la crise sanitaire et ses répercussions industrielles. Une politique tarifaire différenciée en fonction

Une politique tarifaire différenciée en fonction de la localisation des activités de production des entreprises concernées, à laquelle s'ajoute la clause de sauvegarde sur les dispositifs médicaux de la liste en sus, introduite par la loi

Merci

souhaitable d'établir un lien direct entre fixation du prix et implantation des entreprises en France. Bien sûr, nous travaillons pour qu'il y ait des industries de santé en France- c'est un engagement du Gouvernement. Mais cela doit passer par une approche globale et des leviers appropriés, et non pas nécessairement par la loi.

La promotion des biosimilaires réalisée par les industriels qui les produisent relève d'un accompagnement à la recherche d'économies. Le potentiel d'économies supplémentaires

leur vocation est la même : créer des économies pour le système de santé. » Les économies, très bien ; mais cet objectif reste subsidiaire par rapport à l'impératif de protection

au profit de la Caisse nationale de l'assurance maladie, tout comme certains médicaments génériques et orphelins. Pour la plupart sans alternative thérapeutique, ces médicaments sont destinés au traitement de maladies rares et graves. Le législateur a souhaité les exonérer pour

ne bénéficie pas de cette exonération, notamment les médicaments qui ont obtenu une autorisation de mise sur le marché centralisée européenne. Ces médicaments sont pourtant tout aussi essentiels à la couverture des besoins des patients que les médicaments actuellement exonérés.

les indicateurs dont nous disposons en matière de pénurie de médicaments sont au rouge ! Dès 2018, nos collègues Decool et Daudigny avaient tiré la sonnette d'alarme dans un rapport d'information.

d'une actualité brûlante. Je suis évidemment favorable à ce qu'elle fasse l'objet d'un examen approfondi, sur la base des travaux de nos collègues Jean-Pierre Decool et Yves Daudigny. Pour autant,

: en immobilisant la production par site industriel, nous enverrions des signaux délétères à nos différents partenaires commerciaux et prendrions le risque de gripper, en les rigidifiant, les canaux de distribution, dont les situations de crise nous ont montré qu'ils devaient rester souples.

de ce décret est fondamental, car la Commission européenne demande à la France de prouver qu'elle ne lèse pas les autres États membres par une mesure disproportionnée de stockage de médicaments destinés au seul marché national. C'est pourquoi il a été retenu une durée de stocks de deux mois

par décision du directeur général de l'ANSM. Cette liste de médicaments sera régulièrement réévaluée par l'ANSM. Par ailleurs,

pensé à l'origine pour le secteur du médicament. Loin de vider le mécanisme initial de sa substance, il s'agit essentiellement d'une mesure symbolique et cohérente, portant le signal fort de l'ambition de la France en matière d'innovation. de santé (CSIS) doivent ainsi trouver leurs premières traductions un traitement spécifique de la régulation de ce secteur. Actuellement, les dispositifs médicaux se voient appliquer une clause de sauvegarde inadaptée aux spécificités de ce secteur. Le secteur des dispositifs médicaux ne peut être traité avec les mêmes mécanismes budgétaires que ceux qui sont appliqués au médicament, en raison de différences de modèle économique, de processus technologiques et industriels, de tissus d'entreprises, de cycles d'innovation,

sur la liste en sus des dispositifs médicaux les produits et prestations répondant aux deux critères suivants : un niveau d'amélioration du service attendu élevé et une inscription récente sur la liste en sus. Cette exception temporaire permettrait de préserver les nouveaux dispositifs médicaux innovants pouvant nécessiter, dans un premier temps, une diffusion progressive dans les premières années de leur accès au marché, afin de répondre aux besoins d'une population cible qui ne bénéficiait pas auparavant d'une telle innovation.

j'émettrai un avis de sagesse.

Vous souhaitez réduire ou supprimer le périmètre d'application de la clause de sauvegarde. Les dispositifs médicaux présentant un niveau d'amélioration du service attendu majeur à modéré sont la plupart du temps des produits à fort impact budgétaire pour l'assurance maladie.

Elle n'a pas vocation à être le levier principal de la régulation des dépenses. Pour rappel, la clause de sauvegarde est plafonnée à 10 % de l'ensemble du chiffre d'affaires de l'entreprise exploitant un dispositif médical, ce qui doit permettre de rassurer les entreprises sur sa portée. Le Gouvernement ne Le Gouvernement ne souhaite pas revenir sur cette mesure, votée l'année dernière, qui permet une régulation lisible et prévisible. La réduction du périmètre ou l'exclusion

n° 159. Le présent article prévoit la remise au Gouvernement d'un rapport sur les clauses de sauvegarde et l'opportunité de la bioproduction académique afin de rendre les dépenses relatives aux médicaments plus soutenables. Bien que ces deux sujets puissent être indirectement liés, l'objet de ce rapport semble assez mal « ficelé », si vous me permettez l'expression. Le présent amendement vise donc à supprimer cet article.

du rapport visé. Contrairement à ce qui est réalisé dans la production industrielle, des innovations thérapeutiques ciblées et produites ponctuellement sont mises en place en fonction des spécificités des patients, notamment pour les immunothérapies cellulaires. De nombreux laboratoires et centres de recherche investissent massivement dans le développement de ces innovations, qui permettent de réduire les pertes de chances de survie pour de très nombreux patients. Ces innovations particulières ont un coût très important de par leur caractère ciblé et personnalisé. C'est la raison pour laquelle nos collègues députés ont adopté un amendement créant cet article 17 , qui prévoit la remise par le Gouvernement d'un rapport évaluant l'opportunité de produire des biothérapies traitant de pathologies cancéreuses rares pour une utilisation à plus large échelle, ce qui permettrait de réduire le coût que cela représente pour la collectivité. Cette disposition me paraît pour le moins bancale, car elle porte confusion entre les propriétés et capacités des produits traitant des cas ponctuels et spécifiques et ceux qui peuvent être produits industriellement. produits industriellement. Les conditions du suivi de leur qualité et de leur efficacité, et l'assurance d'une équité de traitement pour l'ensemble des patients ne peuvent être garanties si l'on considère ces deux types de produits comme équivalents ou similaires. Le présent amendement vise donc à supprimer l'article 17 . L'urgence de la maîtrise des comptes sociaux ne doit pas nous amener à voter des mesures contre-productives pour les soignants et les patients. Quel

notamment par les virus de l'hépatite C et de l'hépatite B. Cinquante ans après, l'activité contentieuse continue. Alors que l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux peut exercer un recours directement à l'encontre des assureurs des anciens centres de transfusion sanguine sur la base d'un régime de responsabilité sans faute, les organismes d'assurance maladie ne le peuvent pas et sont contraints d'agir contre l'Établissement français du sang, qui se charge d'appeler en garantie les assureurs sans pouvoir bénéficier du même régime de preuves et de responsabilité. Cette situation met à mal les recours des tiers payeurs, qui ne peuvent que difficilement récupérer les débours, et impose à l'Établissement français du sang un rôle d'intermédiaire qui n'est pas efficient.

ans après la création de la sécurité sociale, le Parlement créé une cinquième branche dédiée au soutien à l'autonomie des personnes âgées et des personnes en situation de handicap. Cela fait plus de vingt-cinq ans que les associations attendaient cette réforme. Le Président de la République et vous-même, madame la ministre, avez affirmé que la loi Grand âge et autonomie serait le marqueur

La convergence et la coordination des politiques à destination des personnes âgées dépendantes et des personnes en situation de handicap est bienvenue ; nous l'avons rappelé lors de l'examen de l'article 16. Outre ses missions, le financement de cette cinquième branche est un enjeu.

% d'ici à 2040 ; et parce que nul ne peut se satisfaire des transferts à niveau constant de prise en charge. Les restes à charge pour les personnes âgées dépendantes sont trop élevés, les moyens dont disposent les personnels qui apportent des soins aux aînés ne le sont pas assez, que ce soit à domicile ou en établissement. Par conséquent, les transferts de financement opérés des autres branches vers la nouvelle ne doivent pas cacher le fait que les moyens nouveaux sont dérisoires ne permettront pas, par exemple, de répondre au besoin d'augmentation des effectifs de 25 %- soit la création de 20 000 emplois supplémentaires -pour accorder les soins nécessaires et préserver la dignité des personnes en perte d'autonomie, alors même que les contributions nouvelles que nous avons présentées à l'article 16

un souci de cohérence, a pour objet de supprimer l'organisation du financement de l'ASI au sein de la sécurité sociale, ce financement devant rester à la charge de l'État.

du code de la sécurité sociale : « La sécurité sociale est fondée sur le principe de solidarité nationale. » Il n'y a donc aucun obstacle de principe à ce que l'allocation supplémentaire d'invalidité, qui relève de la solidarité nationale, soit financée par la sécurité sociale. De plus, ce transfert à la sécurité sociale est cohérent, car l'ASI complète la pension d'invalidité, ses bénéficiaires remplissant les mêmes conditions médicales et administratives. Ce transfert permet un meilleur pilotage du risque d'invalidité, en ayant une vision unifiée de ces deux dépenses profondément complémentaires. Pour mettre en oeuvre ce transfert, il est nécessaire de prévoir de nouveaux circuits de financement. Les alinéas que vous souhaitez supprimer sont indispensables au transfert de l'ASI à la sécurité sociale. J'émets donc un avis défavorable sur votre amendement

par l'entreprise pharmaceutique au Comité économique des produits de santé, en intégrant dans la liste des critères de fixation des prix des médicaments, les montants consacrés au financement d'opérations de recherche liées aux produits de santé ainsi que les crédits d'impôt attribués par l'État. Actuellement, les investissements réalisés par les industries, notamment en recherche et développement ainsi qu'en production, peuvent être pris en compte dans la définition du prix. Il faut, selon nous, arrêter de faire payer deux fois le prix au contribuable : une première fois avec le financement public de la recherche et développement dans le domaine biomédical ; une deuxième fois dans le prix final du médicament remboursé par l'assurance maladie. En effet, l'État contribue très largement au développement des médicaments arrivant sur le marché : indirectement, en formant des scientifiques et des chercheurs dans son système d'enseignement supérieur et en investissant dans la recherche publique et le partage des découvertes scientifiques ; et directement, par l'octroi de subventions aux entreprises, telles que le crédit d'impôt recherche-dont nous avons beaucoup parlé-, le crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (CICE) ou encore le crédit d'impôt sur la taxe sur les salaires

Il s'agit d'une gabegie pour les comptes publics : ces 22 milliards s'ajoutent aux 40 milliards du CICE, doublés en 2019. En cumulant le crédit d'impôt et l'allégement patronal, ce sont 142 milliards d'euros qui ont ainsi été accordés aux entreprises au cours du quinquennat sans contrepartie, avec des effets pour le moins discutables. Le bénéfice de ce dispositif n'est en effet pas conditionné à des créations d'emplois, à des investissements écologiques, à des augmentations de salaire ou à des investissements dans la recherche ou la formation. Il y a fort à parier qu'il a plutôt servi à rémunérer les dividendes des actionnaires des grands groupes.

évoque, au mieux, 100 000 emplois créés ou sauvegardés pour 90 milliards d'euros versés. Il est temps de mettre fin à ce gâchis, et il semble absolument inutile d'attendre un an de plus

La parole est à Mme Raymonde Poncet Monge. Nous évoquons ici des exonérations pérennes et non des aides exceptionnelles relatives à la crise sanitaire et à la crise économique que nous traversons.

Il s'agit d'une question de principe d'efficacité des dépenses publiques ; les exonérations du CICE ont démontré leur échec à créer de l'emploi. Nous demandons que les entreprises qui en bénéficient s'engagent à respecter certaines règles

: on va continuer à pleurer sur l'impuissance publique, le déclin de la France, etc. Je ne sais pas si vous vous rendez compte à quel point ça démoralise les Français. Là, il s'agit des conditionnalités des aides publiques.

à une déliquescence de la force d'action de l'État, notamment sur ces questions de répartition des richesses. Il est

connaissant déjà un haut niveau de main-d'oeuvre. Il incite les employeurs à contenir certaines augmentations en bas de l'échelle salariale pour continuer à bénéficier à plein des allégements, conduisant ainsi à ce que certains salariés se trouvent durablement rémunérés au voisinage du SMIC.

et salariale homme-femme. Une très grande majorité de femmes ont des emplois précaires et vivent avec des salaires au-dessous de celui des hommes à qualification

en donnant quelques chiffres. Depuis mercredi dernier, 16h16, les femmes travaillent gratuitement, et ce jusqu'à la fin de l'année, si on tient compte des écarts de salaires entre les femmes et les hommes. Selon les données de l'office statistique de le salaire des Françaises est de 15,5 % inférieur à celui des hommes, contre 15,4 % en 2019. Cela représente, cette année, 39,2 jours ouvrés de travail rémunéré.

professionnelle. Selon une étude du ministère du travail réalisée auprès de 40 000 entreprises françaises de plus de cinquante salariés, seules 6 % des entreprises versent des salaires égaux à leurs employés ; pour les entreprises de 1 000 salariés, seules 1 % d'entre elles sont exemplaires.

L'absence d'accord ou de plan relatif à l'égalité professionnelle fait déjà l'objet d'une sanction financière, qui peut atteindre 1 % des rémunérations versées. Je pense donc que, de ce point de vue, on ne peut être que satisfait.

L'effet serait très hétérogène entre les entreprises : l'effet sur l'emploi viendrait uniquement des entreprises individuelles tandis que les groupes fiscaux les plus bénéficiaires du CICE n'auraient pas systématiquement

L'analyse sectorielle reste peu concluante : les résultats ne sont pas robustes sur l'emploi dans l'industrie tandis que l'effet emploi dans le tertiaire n'est pas directement interprétable comme étant lié au CICE. » Et les effets sont quasi nuls sur les prix

Je voudrais juste appeler l'attention sur le fait qu'il nous paraît curieux que ce montant n'ait pas bougé d'un iota depuis le début de l'examen de ce texte, d'autant que les incertitudes pour 2021

que cet article présente un caractère estimatif et informatif, et non normatif, encore faudrait-il qu'il soit vraiment estimatif et informatif ! L'amendement

qui s'affrontent. D'un côté, les tenants d'une participation plus forte de l'État dans le financement de la sécurité sociale plaident pour le recours à des contributions comme la CSG, qui est payée essentiellement par les salariés et les retraités, parce qu'ils considèrent que la sécurité sociale est finalement l'extension des dépenses sociales de l'État en matière de santé, de famille, de vieillesse, de retraites et de perte d'autonomie. les tenants- dont nous faisons partie -d'une vision dans laquelle la sécurité sociale et l'État ont des rôles complémentaires mais distincts. Cette position fait davantage référence aux racines de la sécurité sociale de 1945 considérons que celle-ci est une caisse commune où l'on partage le produit de la valeur ajoutée, une caisse pour laquelle les employeurs et les travailleurs cotisent selon leurs moyens et reçoivent selon leurs besoins. Ce n'est pas être ringard que de défendre cette sécurité sociale, puisque, contrairement aux start-up et autres entreprises privées qui ont fait faillite, celle-ci a fait la démonstration de sa résistance et de sa capacité d'adaptation durant la pandémie de covid-19. Alors que l'article 19 prévoit la compensation compensation des exonérations de cotisations sociales par l'État, nous rappelons notre opposition au principe même d'exonérations de cotisations sociales. Pour nous, derrière la participation commune de la cotisation sociale, il y a une grande partie du pacte social. Si l'on continue d'exonérer les entreprises de leur contribution à la sécurité sociale et de remettre en cause l'universalité des prestations sociales, le pacte le pacte s'écroulera. Dans la période actuelle, nous pensons qu'il faudrait renforcer ce pacte et le moderniser. C'est le sens de notre amendement n° 962, qui vise à majorer les cotisations des plus hauts salaires, alors que les écarts de salaires ont fortement augmenté ces dernières années. Quel

la majoration serait appliquée. Or, conformément à la jurisprudence du Conseil constitutionnel, la CSG est une imposition de toute nature ; l'ensemble des règles qui la concernent en matière de taux et d'assiette doivent donc être prévues par la loi et ne peuvent être renvoyées à un décret. Le Gouvernement est défavorable à ces deux amendements.

Nous proposons d'instaurer une expérimentation intitulée « Objectif 32 heures », correspondant à une exonération de cotisations pour les salariés qui auront signé un contrat de 32 heures payées L'expérimentation permettra d'étudier l'impact d'une telle mesure sur la productivité de l'entreprise, la santé des salariés, ainsi que son effet sur les besoins en termes de recrutement.

La surmortalité dans ce type d'Ehpad démontre l'urgence d'encadrer les multinationales, qui préfèrent réaliser des profits sur le dos et la santé de nos aînés, plutôt que d'investir pour protéger la santé des résidents et résidentes. Après avoir encouragé le secteur privé

tel esclavage moderne n'est pas acceptable, et on doit sérieusement s'interroger sur la philosophie consistant à gagner de l'argent sur le dos des personnes âgées. notre amendement, nous voulons envoyer un message au Gouvernement comme aux multinationales qui gèrent les résidences pour personnes dépendantes : la santé de nos aînés n'est pas une marchandise comme une autre.

Le coût médian d'une chambre dans un Ehpad privé est de 2 620 euros ; à Paris ou dans les Hauts-de-Seine, ce coût atteint même 3 154 euros. L'accueil n'est pas forcément de meilleure qualité, le taux d'encadrement y est généralement inférieur à celui du secteur public et s'élève, selon la CNSA, à 61 personnes pour 100 résidents, contre 80 % dans les établissements publics les mieux dotés, rattachés à un hôpital. La gestion des maisons de retraite médicalisées est très rentable pour quelques grands groupes privés à but lucratif : Korian, coté en Bourse, a réalisé 15,5 % de marge et un bénéfice de 6 % en 2017. En cinq ans, ce groupe a même doublé le dividende qu'il verse à ses actionnaires. Une maison de retraite est aujourd'hui plus rentable qu'un centre commercial : 4,4 %, contre 4,25 %. Le secteur privé des Ehpad est devenu un produit d'investissement en tant que tel. Les fonds de pension achètent les murs d'une chambre pour 110 000 euros, leur rapportera sans grand risque entre 5 % et 6 % par an, soit davantage qu'une assurance vie, avec un statut fiscal très intéressant de loueur meublé non professionnel. Certains opérateurs privés ont vendu des chambres à des prix surestimés, contraignant les exploitants à baisser les loyers versés aux investisseurs. Les mouvements de fusion et d'acquisition se sont accélérés depuis 2013 dans le secteur privé commercial avec l'émergence de trois mastodontes européens de l'hébergement pour personnes âgées : Korian, Orpéa et DomusVi. La France est le premier investisseur et le premier opérateur européen dans le secteur des résidences pour personnes âgées : vous comprendrez que nous voterons l'amendement de nos collègues.

Nous rendons nous aussi hommage à tous les personnels, quels qu'ils soient. Et lorsque notre collègue défend son amendement, elle parle des groupes qui les emploient, et non des soignants eux-mêmes eux-mêmes ! Bernard Jomier vient de rappeler le taux de rentabilité de ces structures : à ce niveau-là, on pourrait au moins exiger que les personnes qui sont accueillies dans ces établissements

Là où il y a une volonté, il y a un chemin !

conditions, qu'ils maltraitent involontairement les personnes résidant dans les Ehpad, non pas parce qu'ils ne font pas leur travail, mais parce qu'on les oblige à travailler en quelques minutes

très nettement ! La commission a émis un avis défavorable. Elle ne partage pas forcément l'ensemble des orientations figurant dans le rapport, mais a choisi d'amender ce dernier, afin d'affirmer son ambition d'un retour à l'équilibre des comptes sociaux dès que la situation économique le permettra. Quel est l'avis du Gouvernement ?

la maîtrise des comptes sociaux demeure évidemment un impératif, et il est indispensable d'amorcer cette trajectoire de retour à l'équilibre dès que la situation le permettra. À ce titre, le Gouvernement s'est engagé à mettre en place un groupe de travail sur la trajectoire et la gouvernance des finances publiques. Réunissant des experts des finances publiques, notamment des finances sociales, il sera chargé de réfléchir, en particulier, à la fixation de nouvelles ancres de finances publiques à moyen terme. L'objectif est d'assurer la soutenabilité de l'ensemble des finances publiques, y compris des finances sociales. À ce

par branche de l'ensemble des régimes obligatoires de base de la sécurité sociale pour 2020. Il s'agit donc d'un amendement de cohérence permettant d'intégrer, dans l'annexe B portant sur les perspectives pluriannuelles, les modifications votées au niveau des dépenses de l'Ondam et des prévisions de recettes.

le résultat du scrutin. Voici, compte tenu de l'ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du

: La parole est à M. Laurent Burgoa. Depuis plusieurs années, la maîtrise insuffisante des dépenses de soins de ville conduit à une mobilisation des mises en réserve des dépenses des établissements de santé. Les efforts d'efficience de ces établissements sont ainsi absorbés par le dynamisme immodéré des dépenses de soins de ville. L'Ondam exécuté s'avère ainsi éloigné de celui qui a été initialement soumis à l'approbation du Parlement. Comme l'a constaté la Cour des comptes dans son rapport d'octobre 2018 sur l'application des lois de financement de la sécurité sociale, la progression toujours vive des dépenses de soins de ville rend nécessaire l'adoption de mécanismes de régulation propres aux dépenses de ce sous-objectif, mécanismes actuellement inexistants à l'exception des dépenses de médicaments. La Cour des comptes a ainsi réitéré sa recommandation d'instaurer des dispositifs plus complets de suivi et de régulation infra-annuels des dépenses de soins de ville.

Ce mécanisme de gel permettrait de contenir l'accroissement des dépenses et ne pas propager la tension de la maîtrise du sous-objectif des soins de ville aux autres sous-objectifs.

Il existe déjà une procédure d'alerte permettant de suspendre des revalorisations tarifaires, en cas de risque de dépassement de l'enveloppe de soins de ville. Il s'agirait ici d'enclencher cette procédure plus systématiquement. Rien n'assure, toutefois, qu'elle sera effectivement déclenchée. Il serait

Le ministre des solidarités et de la santé a adressé à cette fin une lettre de mission au Haut Conseil pour l'avenir de l'assurance maladie (HCAAM). D'ores et déjà, il est proposé d'associer, dans un cadre commun de discussion stratégique, l'ensemble des acteurs de ville et les représentants des établissements de santé. Ce cadre pourrait être l'Observatoire économique de l'hospitalisation publique et privée, ou le HCAAM lui-même. L'objet de cette discussion associant l'ensemble des acteurs de la santé serait de réfléchir aux priorités médicales de l'Ondam en s'appuyant sur des données épidémiologiques et démographiques. Concrètement, il s'agirait de réfléchir au financement des parcours de soins dans une logique décloisonnée et de proposer des évolutions structurantes. Conformément à l'esprit du Ségur de la santé, cette discussion traduirait la sortie d'une logique comptable de l'Ondam au profit d'une logique médicalisée et de santé. Quel de la commission ? Nous partageons l'objectif de rendre à l'Ondam son rôle d'outil de pilotage stratégique de la dépense de santé.

sur les ressources des établissements de santé publics et privés pour leur donner plus de visibilité. Cette instance serait ici étendue aux professionnels de ville pour prolonger la concertation sur un plus large champ des dépenses de santé, concertation qui devrait évidemment intégrer les enjeux de coordination et les parcours de soins.

Bonne. Cet amendement vise à ce que les mises en réserve prudentielles du PLFSS, elles-mêmes issues de la loi de programmation des finances publiques, portent de manière équilibrée sur les différents sous-objectifs susceptibles de connaître un dépassement, notamment l'enveloppe des soins de ville, au regard de son importance. Le respect de l'Ondam s'inscrit en effet dans une nécessité dont les contraintes doivent être partagées par l'ensemble des sous-objectifs qui le constituent. La Cour des comptes, dans son rapport d'octobre 2018 sur l'application des lois de financement de la sécurité sociale, réitère son appel à « une mise à contribution de l'ensemble des secteurs de l'offre de soins afin d'en assurer le respect, y compris les soins de ville qui en ont été à ce jour exemptés pour l'essentiel Aujourd'hui, alors que le montant des mises en réserve est calculé sur l'ensemble de l'Ondam, seul un mécanisme prudentiel est mis en oeuvre sur les sous-objectifs hospitaliers, soit par des mises en réserve, soit par des annulations de crédits, alourdissant l'effort demandé aux établissements de santé.

apporte une réponse satisfaisante. Il ne me semble pas de bonne gestion que le FIR soit abondé par une enveloppe prudentielle pesant sur un autre sous-objectif. À défaut d'un retrait, la commission a émis un avis défavorable.

à très forte pénibilité, bénéficient d'une faible reconnaissance, notamment salariale, est évidemment une bonne mesure. Mais ces 150 millions d'euros, voire 200 millions

d'amendements pour financer les services d'aide à domicile, plutôt que d'intégrer aux prévisions budgétaires les moyens nécessaires à l'accompagnement du vieillissement de la population. Il serait temps de mettre en oeuvre une politique ambitieuse, qui organise la transformation de notre système d'aide à domicile pour l'adapter au vieillissement, en revalorisant les métiers et salaires, et en accroissant le nombre de professionnels formés. La parole

Il y a un mois, le Gouvernement annonçait vouloir débloquer 200 millions d'euros pour que les aides à domicile qui interviennent chez des personnes âgées ou atteintes de handicap bénéficient d'une hausse de salaire d'environ 15 %. Inséré par l'Assemblée nationale en première lecture, l'article 25 A traduit dans la loi cette volonté. D'une part, il vient reconnaître des professionnels très impliqués dans la crise sanitaire que nous connaissons, d'autre part, il entend favoriser l'attractivité des métiers de l'aide à domicile. Cela, nous le savons, est nécessaire. Ce dispositif consiste en un cofinancement avec les conseils départementaux, effectivement compétents en matière d'aide à domicile. Ainsi, l'enveloppe débloquée par le Gouvernement doit financer la moitié de cette revalorisation, à charge pour le département qui accepterait d'entrer dans cette démarche de financer l'autre moitié. Les crédits seront répartis entre les départements en fonction des dernières données disponibles portant sur le volume total d'activités réalisées par les services. Il s'agit de la même méthode que celle adoptée pour octroyer aux aides à domicile une prime covid exceptionnelle de 1 000 euros par salarié, en vertu d'un dispositif annoncé en août par le Président de la République. Une remarque, pour finir, sur le caractère universel de cette aide : je suis opposée à la discrimination entre privé et public, alors que certains départements, dont le Finistère, ne versent pas la prime covid aux salariés du privé. J'ai rencontré les représentants des entreprises de services à la personne à ce propos et je les ai assurés de mon soutien. Il s'agit de prendre en compte l'ensemble des assistants qui aident les personnes ayant besoin d'une aide à domicile. Nous voterons ce dispositif. Je

qui a été mise en exergue par la crise sanitaire, c'est bien le recrutement et le maintien dans l'emploi des salariés d'intervention et, plus largement, le manque d'attractivité des métiers du domicile. Cette situation obère de plus en plus leur possibilité d'accompagner les personnes en perte d'autonomie.

la revalorisation salariale, fixée par accord collectif national étendu, s'imposera de manière homogène à tous les SAAD de France relevant des mêmes accords de branche. suite, les accords collectifs qui seront agréés seront opposables aux financeurs. Tel qu'il est rédigé, l'article 25 A remet en cause ou, du moins, fragilise largement cette opposabilité en permettant à chaque département de de financer, ou non, le soutien aux professionnels. Cela n'est pas cohérent avec le principe légal de l'agrément national des accords collectifs et de l'opposabilité de ceux-ci. Enfin, cet accord fixe non pas un montant fixe, mais uniquement un plafond : le montant final annuel dépendra des engagements financiers de chaque département. Or ce n'est pas possible puisque ce

concerne le recrutement et le maintien dans l'emploi des salariés d'intervention et, plus largement, le manque d'attractivité des métiers du domicile. Pour y remédier, le dispositif prévu à l'article 25 A se fonde sur les mêmes principes que ceux retenus par le Gouvernement en vue du déploiement du cofinancement de la prime covid pour les SAAD. Or ce dispositif n'est pas adapté aux revalorisations salariales. Aussi, par cet amendement, nous proposons de rationaliser le dispositif gouvernemental en rendant son déploiement uniforme et en précisant que la somme de 200 millions d'euros est un montant fixe réparti entre tous les départements.

Toutefois, plusieurs questions demeurent. D'une part, ce dispositif exclut les intervenants à domicile au titre d'autres aides que la prestation d'assurance vieillesse (CNAV). Des salariés dont la mission et les compétences sont identiques à celles des salariés intervenant au titre de la PCH et de l'APA allouées par les conseils départementaux ne sont, ainsi, pas considérés. D'autre part, un doute demeure, au sein des dispositifs APA et PCH sur l'ouverture de cette enveloppe à l'ensemble des modes d'intervention. En effet, les salariés de l'aide à domicile peuvent certes intervenir selon différentes allocations, mais également selon différents modes d'interventions- gré à gré, accueillant familial, mandataire, etc. Par conséquent, l'accès aux dispositifs doit comprendre l'intégralité des salariés du secteur selon leurs fonctions, et non selon le système d'allocation ou le mode d'intervention. Sans prétendre reconfigurer l'ensemble du financement de l'aide à domicile, cet amendement vise à lever le doute sur ce second point.

la crise de la covid. Or l'aide versée par la CNSA vise à aider les départements dans leur politique d'accompagnement des personnes vulnérables. Elle participe donc d'une politique médico-sociale, et non pas d'une politique de l'emploi

M. Alain Milon. Cet amendement a pour objet d'introduire un dispositif complémentaire compensatoire permettant d'aménager le cadre juridique et financier actuel aux spécificités auxquelles sont confrontés, dans leurs activités de soins, notamment de recours, les établissements d'outre-mer et de Corse, sans alourdir les charges publiques à l'intérieur de l'Ondam hospitalier et sans baisse tarifaire associée.

de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2020 a prévu, dans le même esprit, un rapport sur le financement des établissements hospitaliers dans les collectivités d'outre-mer et de Corse afin d'évaluer les coefficients géographiques liés aux facteurs spécifiques de ces territoires et les différents modes de financement dont ils font l'objet.

Celui-ci craint que les personnels des établissements sociaux et médico-sociaux du champ du handicap ne soient exclus des mesures de revalorisation salariale, malgré les demandes répétées des associations d'élargir les discussions engagées dans le cadre du Ségur de la santé.

Monsieur le président, madame la ministre, les temps ont changé, et ce que l'on vit depuis plusieurs mois a mis en évidence l'importance des professionnels des secteurs social, médico-social et hospitalier.

(Ehpad). La forte mobilisation de ces personnels a conduit effectivement au plan Ségur, qui a permis une augmentation de 183 euros net mensuels. C'est un pas en avant qu'on ne peut que saluer,

et j'espère, madame la ministre, que vous pourrez intervenir afin de mettre fin à ces injustices. Monsieur le président, madame la ministre, pour faire suite aux interventions de mes deux collègues, je voudrais vous alerter sur cet article 25, qui donne une base législative aux compléments de traitement indiciaire. Vous parlez d'exclusion ; or ce texte exclut de son champ d'application les agents des groupements d'intérêt public (GIP) qui sont fonctionnaires hospitaliers et qui ont une activité dans le domaine sanitaire. Il prévoit, en revanche, expressément que les agents mis à disposition ou les agents contractuels des groupements de coopération sanitaire (GCS) bénéficient de cette mesure. Cette exclusion des GIP crée une différence de traitement entre les agents publics

La mutualisation au sein des GIP d'activités de logistique hospitalière s'est développée, soutenue d'ailleurs par l'État, afin d'améliorer l'efficience du dispositif hospitalier. dispositif hospitalier. Pour prendre l'exemple de mon département des Côtes-d'Armor, deux structures interhospitalières traitent le linge de l'ensemble des établissements membres du groupement hospitalier de territoire (GHT) d'Armor et emploient des fonctionnaires hospitaliers. Les agents fonctionnaires mis à disposition de l'un, organisé sous forme de GCS, bénéficient de la mesure de revalorisation, tandis que les agents fonctionnaires mis à disposition de l'autre, organisé sous forme de GIP, n'en bénéficient pas. Il s'agit, selon nous, d'une injustice incompréhensible incompréhensible pour les agents concernés. Ils ont le sentiment que leur métier est méprisé, non reconnu, alors qu'ils contribuent comme les autres agents hospitaliers à la lutte contre la covid. Ils sont les invisibles de la chaîne, pourtant essentiels à la bonne marche de l'hôpital.

Le Ségur de la santé aurait pu être l'occasion de le reconnaître à sa juste valeur : force est de constater que ce n'est pas le cas. De nombreux professionnels ont été oubliés. En effet, ce sont près de 40 000 agents de la fonction publique hospitalière qui ne bénéficieront pas de la revalorisation de 183 euros mensuels net. Ainsi, les personnels des établissements sociaux et médico-sociaux en sont exclus. Pourtant, les aides médico-psychologiques, les aides-soignants, les personnels affectés au soutien gérontologique ou à l'accompagnement du handicap, comme les autres professions de ces établissements, ont été en première ligne dès le début de l'épidémie de covid-19. Ils s'y trouvent encore aujourd'hui. Cette différence de traitement inspire un sentiment d'injustice auquel il faut répondre. Les élus du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain avaient proposé un amendement

Mélot, sur l'article. Les accords du Ségur de la santé ont été signés le 13 juillet dernier par le Gouvernement et une majorité d'organisations syndicales. à 1,5 million de professionnels. C'est une reconnaissance méritée de leur dévouement au service des patients et résidents des divers établissements. À cet égard, je salue l'action du Gouvernement : elle permettra de rendre les métiers d'infirmier et d'aide-soignant plus attractifs.

dénombrait 2,5 millions de personnes dépendantes : il en comptera 4,5 millions en 2050. Ces personnes souhaitent, et souhaiteront, rester à domicile le plus longtemps possible.

Merci

ainsi que des agents des établissements et des services sociaux et médico-sociaux, dans le champ d'application du décret du 19 septembre 2020, qui a fait suite aux négociations du Ségur de la santé. Chaque jour, ces professionnels accompagnent et soutiennent à domicile des personnes âgées ou en situation de handicap. Leur travail est indispensable et leur engagement exemplaire, notamment dans le contexte sanitaire que nous connaissons actuellement.

des groupements de coopération sanitaire et des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes de la fonction publique hospitalière. Pour davantage Pour davantage d'équité, il faut envisager l'extension du champ d'application de ce décret par une connaissance accrue de la situation, grâce à un rapport d'information projetant l'intégration des agents des Ssiad, ainsi que des agents des établissements et des services sociaux et médico-sociaux ! La parole

Le Ségur, cela fut aussi 90 participants, 100 réunions bilatérales, 200 réunions territoriales, 118 407 participants qui ont remis des avis en ligne.

de retraite créé en 1960 pour inciter les professionnels de santé libéraux à être conventionnés. Il vient compenser les honoraires contraints par la convention avec l'assurance maladie par le biais d'une participation de l'assurance maladie aux cotisations de retraite.

Pour les auxiliaires médicaux libéraux, l'assurance maladie prend ainsi en charge les deux tiers de la part forfaitaire de la cotisation annuelle et 60 % de la cotisation proportionnelle aux revenus. Des négociations pluriprofessionnelles avaient été lancées à l'occasion des débats sur la réforme du système de retraite, afin d'offrir une solution à la hausse des cotisations ainsi engendrée. Cet amendement d'appel vise à rendre possible la réouverture de ces négociations pluriprofessionnelles, brutalement interrompues du fait de la crise sanitaire. dans la lettre de mission du nouveau directeur général de la CNAM, le ministre des solidarités et de la santé a souligné la mobilisation exceptionnelle des professionnels de santé, qui a permis de faire face à la première vague de l'épidémie de covid-19. Certes, le PLFSS pour 2021 met en oeuvre les engagements du Ségur de la santé liés à la revalorisation des carrières des personnels non médicaux dans les établissements de santé et les Ehpad. il est également temps de saluer la large participation des praticiens de santé libéraux à la continuité des soins sur l'ensemble du territoire auprès de personnes isolées et fragilisées dans ce contexte sanitaire. Il faut donc inscrire l'ASV au coeur des futures négociations conventionnelles pluriprofessionnelles afin de renforcer les engagements réciproques entre les professionnels de santé et l'assurance maladie. Quel est l'avis de

En effet, près de la moitié du plan de 100 milliards d'euros repose sur les engagements de l'Union européenne. Mais les États partisans de l'austérité sont toujours aux commandes, malgré la remise en cause permanente du capitalisme et particulièrement du libéralisme financiarisé. Nous n'accepterons pas davantage l'argent de l'Union européenne soumis, en contrepartie, à des mesures régressives comme la réforme des retraites ou la suppression de postes de fonctionnaires. L'article 26 est justement le bras armé du Gouvernement pour imposer des plans d'austérité dans les hôpitaux qui bénéficieront de la reprise partielle de leur dette.

une politique alternative : l'État doit assumer intégralement la reprise de la dette des hôpitaux et profiter des taux d'intérêt négatifs

ne permettront pas de faire face à l'état d'obsolescence et de vétusté dans lequel se trouvent de nombreux établissements de santé dans notre pays. Les capacités d'autofinancement sont dégradées, voire négatives, pour plus du tiers de nos hôpitaux.

ma chère collègue. Par lettre en date du 12 novembre 2020, M. Bruno Retailleau, président du groupe Les Républicains, demande le retrait de l'ordre du jour du mardi 17 novembre 2020 de la proposition de loi tendant à adapter les règles de passation des marchés publics locaux, conséquence de la crise sanitaire. Acte est donné de cette demande. J'informe le Sénat que des candidatures pour siéger au sein de la commission mixte paritaire chargée d'élaborer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif au retour de biens culturels à la République du Bénin et à la République du Sénégal